En particulier, il est prévu que le montant de la DGF ne puisse diminuer au-delà de celui que percevaient les communes fondatrices l'année de fusion. À l'issue de cette période, les dotations perçues par les collectivités locales sont déterminées dans les conditions de droit commun, en mobilisant notamment leur potentiel fiscal. Or plusieurs phénomènes peuvent conduire la commune nouvelle à observer une baisse des dotations qu'elle perçoit. Tout d'abord, son potentiel fiscal peut avoir augmenté lorsqu'elle a rejoint dans le courant de la fusion un EPCI à fiscalité

structure. Ensuite, la population de la commune nouvelle peut aussi être plus importante, et c'est souvent le cas, que celle des communes fondatrices, si bien qu'elle se compare désormais à d'autres strates démographiques. Elle peut dès lors perdre son éligibilité à certaines dotations, comme la dotation de solidarité rurale. rurale. Parmi les propositions formulées par les différents amendements, la plupart ont pour objet, d'une manière ou d'une autre, de prolonger les garanties existantes ou d'en introduire de nouvelles. Comme vous le savez, nous sommes plutôt défavorables à ces propositions. En effet, d'une part, dans une enveloppe fermée de DGF, les garanties sont toujours financées par les autres communes, ce qui ne se justifie pas nécessairement

Il pourrait donc se poser des problèmes d'équité par rapport aux autres communes qui sont dans le même cas. Toutefois, nous comprenons l'inquiétude que suscite pour nombre de communes nouvelles une sortie sèche de ces garanties. Aussi, nous pensons que l'amendement n° II-438 rectifié de Mme Gatel peut constituer un point de départ. Il vise à introduire un dispositif de sortie en sifflet sur quatre ans en cas de perte d'éligibilité d'une commune nouvelle à la dotation de solidarité rurale ou à la dotation nationale de péréquation. Un tel mécanisme nous semble excessif, mais nous en comprenons l'intention. Nous proposerons donc à Mme Gatel une donc à Mme Gatel une rectification de son amendement tendant à prévoir que, lorsqu'une commune nouvelle perd son éligibilité à la DSR ou à la DNP, elle bénéficie, l'année suivant la fin du pacte de stabilité, d'un versement égal à 50 % des ressources perçues l'année précédente.

! Il se trouve que, en 2018, le comité des finances locales a voulu travailler sur la réduction des inégalités de dotations entre catégories d'intercommunalités, à savoir les métropoles, les communautés urbaines,

? Françoise Gatel, Élisabeth Doineau et Agnès Canayer ont déposé des amendements relatifs au régime des communes nouvelles.

toutes les communes d'un même EPCI ne sont plus tenues d'adhérer à une nouvelle intercommunalité ; elles conservent alors les dotations de l'ancien EPCI au niveau communal. Je ne suis pas favorable à la modification de ces règles, qui constituent à mes yeux un point d'équilibre entre les avantages accordés aux communes nouvelles et le principe d'égalité de traitement dans le calcul de la DGF. de souligner que les règles actuelles bénéficient largement aux communes nouvelles. Elles reçoivent en moyenne 220 euros par habitant

les amendements visant à créer une garantie définitive du montant de la DGF ne sont pas envisageables, ne serait-ce que pour des raisons constitutionnelles. dans un instant, vise pour sa part à lisser dans le temps la sortie du pacte de stabilité. Entendons-nous bien : il s'agit en fait d'une garantie de sortie de la garantie de sortie de la garantie de sortie ! À l'issue des trois années de garantie, une commune nouvelle qui verrait sa DGF baisser pourrait bénéficier de quatre nouvelles années de garantie, dégressives cette fois.

Mon silence valait réponse.

La Cour des comptes a relevé dans son rapport sur les finances locales de 2017 que les dotations de péréquation verticale des communes des DOM, logées dans la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (Dacom), étaient inférieures de 100 millions d'euros

les insuffisances de la péréquation nationale à l'égard des outre-mer et s'est engagé à un rattrapage à hauteur de 85 millions d'euros. Le PLF pour 2020 a acté un rattrapage de la Dacom de 55 millions d'euros

qu'il fallait accélérer ce rattrapage en réduisant le délai d'un an pour tenir compte de la crise économique, ce qui n'est pas suffisant. Le présent amendement vise à réaliser l'intégralité du rattrapage restant dès l'année 2021.

Le PLF pour 2020 a instauré une majoration démographique de la dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer au profit des chefs-lieux de département et d'arrondissement de plus de 10 000 habitants, afin de répondre aux enjeux de centralité des villes capitales d'outre-mer. Concernant les chefs-lieux d'arrondissement, la mesure ciblait plus particulièrement Pointe-à-Pitre et Saint-Laurent-du-Maroni, capitale de l'ouest guyanais. Il se trouve que cette majoration démographique bénéficie surtout aux chefs-lieux d'arrondissement les plus peuplés. peuplés. Ce critère démographique a moins d'impact sur les capitales guadeloupéennes, qui sont peu peuplées- 13 000 habitants en moyenne pour une population régionale de 420 000 habitants -, alors que ces dernières supportent des charges de centralité hors normes : 803 euros par habitant pour Basse-Terre, plus de 500 euros par habitant pour Pointe-à-Pitre, contre 133 euros par habitant pour les autres villes capitales, selon une étude de la DGOM en De plus, du fait de son déclin démographique, Basse-Terre risque de passer sous la barre des 10 000 habitants dans les prochaines années et ainsi perdre le bénéfice de cette majoration. Le présent amendement vise donc à sécuriser l'éligibilité de Basse-Terre à cette majoration, tout en renforçant la majoration démographique de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre et en diminuant celle des chefs-lieux d'arrondissement les plus peuplés, dont le niveau de charges de centralité est moins élevé.

Comme vient de le dire M. le rapporteur spécial, il s'agit d'une réforme qui a été négociée avec les élus d'outre-mer, l'année dernière. Elle touche aux modalités de répartition d'une dotation qui n'a été répartie qu'une seule fois en 2020.

encore moins la légitimité d'une telle péréquation horizontale. Aujourd'hui, 1 milliard d'euros est redistribué en France, essentiellement de régions industrielles et très dynamiques économiquement

ne sont donc plus du tout les mêmes, d'où l'incompréhension qui naît de la mise en oeuvre du FPIC sur les territoires. Cet amendement a pour objet de revenir sur les critères issus de l'article 78 de la loi de finances pour 2010, de manière qu'ils ne soient plus pris en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé par habitant.

ne me semble pas justifiée, puisque ces montants demeurent une ressource ou une moindre ressource pour les collectivités locales. Ainsi, à recette fiscale équivalente, un ensemble intercommunal qui perçoit un reversement au titre du FNGIR est

En plus, on a un débat moralisateur : ce seraient les riches qui ne voudraient pas donner aux pauvres. Je pense que, dans cet hémicycle, il y a trop d'intelligence pour qu'on caricature les choses.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à neutraliser les effets du transfert d'une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal de ces collectivités Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a bien été réduit de la part de CVAE transférée à la région, mais, comme cette contribution représente une plus forte proportion des ressources dans les départements riches, ces derniers a été plus fortement réduit que celui des départements dits pauvres, ce qui avantage les départements riches dans les calculs de péréquation. Nous proposons de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale et, à l'inverse, de considérer les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L'objectif est de corriger l'effet contre-péréquateur du transfert de CVAE. Je précise que ce type de mécanisme de correction existe déjà au sein du bloc communal, pour tenir compte des attributions de compensation des EPCI en fiscalité professionnelle unique.

vise à faire respecter pleinement les termes de l'accord de partenariat conclu entre l'État et les régions le 28 septembre dernier. Nous sommes pour

vise ainsi à supprimer le dispositif transitoire prévu à l'article 58 dans sa rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. En second lieu, l'amendement tend à supprimer les dispositions du même article qui préfigurent les contours du futur système de péréquation des ressources régionales, qui doit se concrétiser en 2022. Vos rapporteurs spéciaux partagent l'objectif d'un renforcement de la résilience financière des régions, qui passe par un effort accru en faveur de la péréquation horizontale de leurs ressources, aujourd'hui insuffisante. Ils se félicitent donc que l'accord prévoie l'engagement de négociations entre l'État et les régions pour une rénovation du système de péréquation. Néanmoins, la méthode retenue interroge, dans mesure où elle préempte largement l'issue des négociations en fixant, dès le projet de loi de finances pour 2021, le volume des ressources mises en répartition- 1 En outre, en opérant un renvoi général au décret, le dispositif proposé ne permet pas au législateur de se prononcer sur des modalités de répartition des ressources du fonds, en particulier sur la définition des critères de ressources et de charges. Nous invitons le Sénat à supprimer ces dispositions dans l'attente

Instauré consécutivement à la réforme de la taxe professionnelle, ce fonds est calculé pour chacune des régions : lorsque le pourcentage de croissance excède la moyenne, un écrêtement est opéré qui ramène de fait la région considérée dans la moyenne le produit ainsi collecté est servi aux régions en configuration inverse, elles-mêmes renvoyées à la moyenne. Ce mode opératoire aboutit à homogénéiser le taux de croissance des ressources fiscales venues en remplacement de la part régionale de taxe Les écarts constatés en 2011, l'année de référence, sont donc figés, ce qui prive les territoires bénéficiant d'une croissance économique de l'intégralité du bonus fiscal induit. C'est la raison pour laquelle le code général des collectivités territoriales exonère les régions d'outre-mer de ce prélèvement. Dans ce prolongement, il est peu compréhensible que la Corse ne bénéficie pas, elle aussi, de cette dispense de prélèvement, compte tenu de son indice de ressources fiscales, de loin le plus bas de la métropole.

Dans le contexte actuel de crises sanitaire et économique et compte tenu de la baisse sensible de la fréquentation touristique dans l'île, il paraît injuste et pénalisant que la Corse contribue à ce fonds du fait qu'elle dispose d'une ressource fiscale évoluant plus vite que la moyenne. faut considérer que cette ressource est nettement plus faible que dans les autres régions. Un rattrapage économique a été accompli ces dernières années, mais la crise de la covid-19 donne un coup d'arrêt à ce relatif dynamisme économique, lié au secteur du tourisme et aux activités qui en découlaient.

révision du système de péréquation entre les régions, rappelle que des discussions ont déjà été engagées à cet effet et précise : « L'État et les régions s'engagent, dans le PLF 2021, à finaliser les dispositifs correspondants à l'été 2021, pour une traduction législative dans le PLF 2022.

je vous le dis très honnêtement. Quand des accords sont conclus, je ne suis pas du genre à ne pas les tenir : vous pourrez demander aux départements comment ça s'est passé la semaine dernière ...

qui minore davantage le potentiel fiscal des départements riches, fortement dotés en CVAE, que celui des départements pauvres, moins bien pourvus. Ce constat doit être nuancé. En effet, la perte d'une part de CVAE, même compensée par une attribution de compensation, correspond bien à une baisse du potentiel fiscal, qu'il me paraît difficile de neutraliser, comme si le transfert n'avait jamais eu lieu. En pratique, l'éligibilité au mécanisme de péréquation en 2018, 2019 et 2020 s'est révélée très stable. La question était plus prégnante pour les régions, puisque le fonctionnement de leur fonds de péréquation a pour effet de démultiplier les contributions en cas de progression de leur panier de ressources. Ce point a été identifié et traité, en liaison avec l'ARF, dans 2018. Je ne suis donc pas convaincue qu'il faille modifier le calcul du potentiel fiscal des départements pour neutraliser les effets, au demeurant limités, du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2018. les montants de ces compensations ont été déterminés en fonction d'échanges entre les départements et les régions et d'accords entre eux. Je verrais un problème important à modifier les conditions de ces accords négociés entre collectivités territoriales.

est astreinte au même régime de répartition de prélèvements ou de reversements que les autres régions métropolitaines. Je ne vois pas de raison d'introduire une dérogation pour 2021. je vous remercie

sur les petites communes à dimension touristique, d'autant plus lourdes dans le contexte économique incertain auquel elles font face. Alors que tout doit être fait pour faciliter l'investissement dans le cadre de la relance économique, les communes touristiques, notamment les communes supports de stations de montagne, sont fortement contributrices au FPIC, du fait de leurs ressources fiscales plus élevées que celles des autres communes de même strate de population. Mais ce calcul ne tient pas compte des charges et dépenses spécifiques qu'elles supportent, en termes d'aménagement, d'investissement et de sécurité pour les vacanciers. Je pense à l'assainissement, aux routes, aux structures : tout est surdimensionné et présente des coûts de mise en oeuvre supérieurs en terrain de montagne. Ce déséquilibre fragilise la situation budgétaire de ces communes et diminue leur capacité d'investissement et surtout de maintien à niveau de leur outil économique. Dans le contexte actuel, une telle diminution serait préjudiciable pour le secteur touristique français, qui a plus que jamais besoin de soutien.

Afin de limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, comptant moins de 10 000 habitants. En effet, le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités en 2019 fait apparaître un véritable effet de seuil : au-dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes.

qui vise à avantager les communes de montagne dans le calcul des dotations. En effet, plusieurs de ces communes considèrent que les différents dispositifs de péréquation ne prennent pas suffisamment en compte les charges auxquelles elles sont exposées. Le nombre de résidences secondaires constituerait à cet égard un moyen d'approcher la réalité de ces charges. Il s'agit d'ailleurs d'une approche plutôt cohérente, puisque le nombre de touristes est bien corrélé au nombre de résidences secondaires. Toutefois, je tiens à rappeler que divers mécanismes conduisent déjà à majorer la population DGF en fonction du nombre de résidences secondaires. L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la population DGF est majorée d'un habitant par résidence secondaire. L'article L. 2334-7 du même code prévoit que la population DGF est majorée de 0,5 habitant par résidence secondaire lorsque la population est inférieure à 3 500 habitants, lorsque le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de la strate démographique démographique et lorsque la population des résidences secondaires représente plus de 30 % de la population DGF après application de la majoration de droit commun. Ainsi, si les mécanismes de péréquation ne tiennent pas ne tiennent pas suffisamment compte des charges qui pèsent sur les communes de montagne, le levier de la majoration de la population DGF en fonction du nombre de résidences secondaires semble avoir atteint ses limites. Jusqu'à quel point faudrait-il encore le majorer ? On ne peut pas majorer la population DGF d'un demi-habitant par Par ailleurs, l'adoption de cet amendement entraînerait nécessairement des effets de bord, alors que l'amélioration de la situation des communes de montagne n'est pas certaine. Enfin, je rappelle que les communes disposant de nombreuses résidences secondaires sont celles qui, paradoxalement, vont subir le moins fortement le contrecoup de la réforme de la taxe d'habitation. En effet, elles continueront à exercer un pouvoir de taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans ce contexte, mes chers collègues, vous comprendrez que la commission des finances ait rendu un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements,

vise à corriger une profonde injustice entre communes rurales et communes urbaines. Je suis sûr que le secrétaire d'État ne pourra que me rejoindre, montrant ainsi l'utilité que nous ayons enfin un secrétaire d'État chargé de la ruralité.

montrent que ces différences de charges selon la taille des communes sont largement sous-évaluées pour les petites communes et surévaluées pour les grandes communes. Cet amendement vise donc, non pas à supprimer totalement la différence

la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitant par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %. Toutefois, se fonder sur le potentiel fiscal se révèle pénalisant pour les communes touristiques qui bénéficient de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique. Néanmoins, ces mêmes communes supportent des charges touristiques bien plus élevées, créant un déséquilibre en leur défaveur.

Il est également précisé que le seuil de 3 500 habitants retenu s'applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a en effet trouvé des difficultés à s'appliquer, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n'en ayant pas bénéficié en raison d'une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué. Or retenir la population DGF au lieu de la population municipale pour appliquer le seuil paraît incohérent avec l'objectif même de cette majoration. ce dispositif devait permettre aux petites communes de bénéficier d'une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire afin de prendre en compte leurs charges touristiques. je vous remercie

Aujourd'hui, du fait de la montée de l'intercommunalité, ce paysage a complètement changé. De plus, nos concitoyens nous font remarquer que, désormais, quelle que soit la taille de la commune dans laquelle ils habitent, ils sont souvent soumis au même niveau d'imposition.

alors même qu'elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, parfois avec un potentiel fiscal quinze fois supérieur au seuil d'écrêtement. Pour remédier

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement a pour objet d'indiquer que, pour les communes dont le potentiel financier est supérieur à deux fois la moyenne nationale, le montant de l'écrêtement peut excéder celui de celui de la dotation forfaitaire. En d'autres termes, ce mécanisme conduira à faire financer la péréquation horizontale en partie par des prélèvements sur les recettes de fiscalité des communes les plus riches. On observera qu'en l'absence d'une participation plus importante de l'État, une augmentation de la DGF, cette solution garantira une hausse des dotations de péréquation.

des collectivités, imputée à titre principal sur la DGF et à titre secondaire sur la fiscalité. La dotation forfaitaire est un vecteur technique de contribution, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

ni cohérent de prélever une part de la fiscalité de certaines communes pour financer le dynamisme des dotations de péréquation, les garanties de DGF sur les communes nouvelles et d'autres mesures de ce type. En outre, votre amendement ne tourne pas

Comme vous le savez, la part forfaitaire de la DGF tient compte de la variation de la population de chacune de ces communes, avalisée par l'Insee au début de chaque année. À l'heure actuelle, les communes perçoivent 64 euros par habitant supplémentaire lorsqu'elles ont moins de 500 habitants et 128 euros si leur population dépasse 200 000 habitants. Que se passe-t-il entre les deux ? Une formule mathématique attribue un coefficient à chaque commune, d'autant plus proche de deux que sa population approche 200 000 habitants. Je vous épargnerai cette formule où un nombre à huit chiffres après la virgule côtoie un logarithme décimal.

des charges de centralité et où il est nécessaire d'accompagner le dynamisme de nos territoires ruraux jusqu'à la plus petite commune, ce dispositif n'a plus lieu de perdurer. Aussi, je vous propose de ramener l'écart, qui est actuellement du simple au double, à un rapport de 1 à 1,6. 1,6. La dotation se calculera encore avec un coefficient logarithmique, mais par une formule beaucoup plus simple. Si cet amendement est adopté, les communes de moins de 1 000 habitants seront traitées comme celles qui ont exactement 1 000 habitants.

Cet amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dite « bourg-centre notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et que la crise économique et sociale induite par l'épidémie de covid-19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinent d'encourager les communes rurales, qui prennent leur part de la solidarité nationale, en produisant de tels logements. Le Gouvernement souhaite que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie.

La première fraction de la DSR est actuellement attribuée aux communes rurales en fonction des critères de proximité avec une agglomération, de population et de potentiel financier. Introduire une conditionnalité supplémentaire dans l'attribution de la DSR pour l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants ne semble pas être le moyen le plus efficace pour favoriser le respect des seuils d'obligations de logements sociaux.

Par ailleurs, la DSR n'a pas vocation à être un outil incitatif, car il s'agit simplement d'une dotation de péréquation. D'autres instruments pourraient être plus utilement mobilisés tout en ayant un impact moins négatif sur les plus petites communes,

l'ampleur des travaux que le conseil départemental doit affronter après la catastrophe récemment survenue : ils sont évalués à 850 millions d'euros pour les voiries et ouvrages d'art.

? Monsieur le sénateur Arnaud Bazin, je confirme ce que vient de dire le rapporteur spécial. Sur le plan de la forme, il s'agit sûrement d'un amendement d'appel, car il n'a pas de portée normative. Sur le fond, le Gouvernement partage votre volonté de soutenir financièrement le département des Alpes-Maritimes. Néanmoins, agir sur la péréquation n'est pas un bon vecteur pour résoudre des situations liées à des catastrophes naturelles. Ce genre d'événement exceptionnel appelle nécessairement des réponses ciblées, adaptées aux circonstances précises du sinistre.

Je tiens à vous préciser que l'État a d'ores et déjà annoncé qu'il saurait pleinement assumer ses responsabilités et apporter un soutien important aux collectivités concernées.

Enfin, la DGF étant calculée avec les données de l'année-1, cette garantie ne s'appliquerait qu'à compter de 2022, année où la DGF sera calculée avec le nouveau panier de recettes fiscales ? Mon cher collègue, votre amendement vise à ce que la DGF par habitant des EPCI ne puisse plus baisser d'une année sur l'autre. À enveloppe constante, des garanties de cette nature se font nécessairement au détriment des communes dont le potentiel fiscal diminue

Le Gouvernement devait rendre un premier rapport en application du XI de l'article 250 de la loi de finances pour 2020, mais celui-ci n'a toujours pas été remis, ce qui nous empêche-

en fonction croissante de la population des communes et des ensembles intercommunaux, sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes et du FPIC. Si ce rapport de 2019 a conclu à la pertinence de l'outil et à son efficacité dans l'appréhension du niveau de charges des collectivités au regard de leur population, il souligne néanmoins la nécessité d'approfondir la réflexion sur les bornes au sein desquelles ce coefficient évolue et, par incidence, sur le niveau de variation de celui-ci.

est l'avis de la commission ? Il s'agit d'une demande de rapport sur les charges exceptionnelles assumées et les recettes perçues par les collectivités locales.

soutenir les secteurs de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics. Dans le cadre du droit existant, conformément au code général des collectivités territoriales, la DETR est calculée en tenant compte de la population de l'ensemble des communes qui sont situées

propose une DETR stable, à hauteur de 1,046 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 888 millions d'euros en crédits de paiement. Les projets d'investissement sont

départements. Il importerait donc d'encadrer plus strictement les variations de la DETR accordée à chaque département pour relier la dynamique de la dotation aux évolutions démographiques. L'amendement n°

en prenant davantage en compte la densité des communes. Elle a montré que cela conduirait à rendre inéligibles 3 304 communes qui ont toujours pu bénéficier de la DETR jusqu'à présent. Je suis en accord avec vous, mon cher collègue, sur le fait que cette réforme serait nécessaire pour redonner plus de poids aux communes rurales, mais elle ne peut être menée qu'après une négociation approfondie pour limiter au maximum le nombre

le dis en toute tranquillité. Écoutez-moi bien : nous ferons passer en fin de soirée la liste des 3 304 communes exclues de

Je trouve que ce serait une leçon pour nous tous. Je vous le dis très gentiment, monsieur Belin : j'ai beaucoup de respect pour nos collègues de l'Assemblée nationale, surtout lorsqu'ils travaillent en intergroupe et qu'ils essayent de trouver des solutions intelligentes en faisant des simulations.

chaque fois qu'il y a une réforme de la fiscalité locale, nous exprimons le souhait qu'elle soit indépendante du débat budgétaire : nos communes méritent mieux que d'être la variable d'ajustement du budget. Il ne faut pas vous étonner si vous avez autant d'amendements, puisque vous refusez systématiquement la réforme de fond en la renvoyant à des jours meilleurs. Nous n'avons pas d'autre solution que de déposer ces amendements. Nous sommes bien conscients qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils comportent des risques. Pour autant, je vais voter cet amendement, simplement pour manifester ma mauvaise humeur. Il est peut-être temps que le Gouvernement comprenne que la réforme de la fiscalité n'est pas la variable d'ajustement du budget et qu'il est temps de se mettre au boulot

sont tous éligibles, sauf s'ils cumulent deux conditions : avoir une commune centre de plus de 20 000 habitants et avoir une densité de population par habitant supérieure à 150 habitants par kilomètre carré.

citée par le rapporteur spécial Claude Raynal a été instaurée, mission parlementaire qui d'ailleurs, que je sache, est venue rencontrer les principaux responsables du Sénat pour présenter ses travaux.

perçue par les EPCI aux projets que ces derniers réalisent sur le territoire de leurs communes membres qui sont elles-mêmes éligibles à la DETR. On ne modifie pas le champ des EPCI et, donc, aucun ne se trouve exclu du dispositif. On ne modifie pas non plus le registre des communes éligibles,

pilote ». Les critères d'éligibilité de la DETR ne cessent d'évoluer depuis des années pour, que l'on subventionne des communes de plus de 30 000 habitants l'EPCI dont elles sont membres- je ne citerai aucun nom, bien entendu, pour éviter toute stigmatisation.

dans les départements de métropole, comme c'est déjà le cas dans les départements d'outre-mer, et, d'autre part, à rehausser au-delà de 3 500 habitants le seuil d'exigibilité

Le mieux étant l'ennemi du bien, il est alors tout à fait possible que les crédits soumis à cette double condition et ainsi fléchés ne soient jamais consommés. Par conséquent,

à l'investissement des collectivités territoriales de l'État et, d'autre part, de mieux associer les élus locaux aux décisions d'attribution de subventions. À l'exception notable de la DETR, nous en avons parlé à de nombreuses reprises, les élus locaux ne sont pas nécessairement informés ou associés aux décisions d'octroi des subventions. Je précise que cette

Merci,

Cet amendement vise à inclure, sans en augmenter l'enveloppe, les investissements touristiques dans les catégories d'opérations éligibles à la DSIL. Pour mémoire, les communes touristiques contribuent aux millions d'emplois directs et indirects liés au secteur économique du tourisme,

Il est nécessaire de conserver sur le long terme cette attractivité, cet avantage compétitif, en apportant notre soutien aux communes touristiques- ou plutôt « communes entreprises

liste : s'y ajoutent la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ; le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; enfin, la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires

n° II-580 rectifié. Cet amendement vise à donner au préfet de département le rôle d'attribuer les subventions au titre de la DSIL, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région. Par ailleurs, il tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la DETR et de la part départementale de la DSIL. Cette commission serait modelée sur l'actuelle commission DETR, mais ses compétences seraient renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention adressée au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées. En résumé, il s'agit d'un amendement de simplification. Aujourd'hui, le préfet de région demande au préfet de département, qui lui-même se tourne vers les sous-préfets d'arrondissement, quels sont les dossiers éligibles à la DSIL. Ensuite, ces dossiers remontent jusqu'au préfet de région.

Pourquoi l'une pourrait-elle se dispenser d'une commission d'élus et l'autre non ? Nous proposons donc de nous inspirer du modèle de la commission DETR pour créer une commission DSIL composée de parlementaires et d'élus locaux,

de proximité. À nos yeux, la complémentarité des dispositifs doit être préservée

de cofinancement par les collectivités, fixé à 20 %, pour les projets recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique provenant de la mission « Plan de relance ». Nous souhaitons introduire un dispositif complémentaire visant des projets plus divers. Par cet amendement, nous proposons d'abaisser également, de manière temporaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, le seuil de participation minimale des petites communes aux projets d'investissement à 10 % au lieu de 20 %. de 20 %. Cette mesure concernerait les communes de moins de 2 000 habitants, principalement rurales, afin que celles-ci puissent participer à la relance de l'économie et accompagner les entreprises locales. Ces communes,

! Le présent amendement tend en réalité à étendre le nombre de bénéficiaires de la DPEL y compris, et c'est là le problème, pour les petites communes rurales les plus riches.

le reste pouvant être réparti selon des critères librement choisis, à la double condition que ceux-ci ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires à 35 % et qu'ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les C'est pourquoi cet amendement vise à assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35 %, et le caractère péréquateur des critères librement choisis. Cela donnerait un peu plus de libertés aux élus locaux dans la répartition des enveloppes et permettrait d'éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.

la vocation est d'apporter une aide financière aux communes afin d'assurer l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux dangereux et qui en sont, par exemple, expulsés à la suite d'un arrêté de péril.

Depuis lors, le Sénat a délibéré sur la première partie de cette loi de finances et a, notamment, voté des mécanismes de compensation de la perte de CVAE pour l'ensemble des EPCI. La raison qui avait poussé les députés à ne

puisque la part des fonds de compensation des charges territoriales et de la dotation de soutien à l'investissement territorial correspondant au produit de la CFE serait neutralisée pendant cette période.

! Je ne pense pas qu'il faille, si vous me passez l'expression, mettre la charrue avant les boeufs en tranchant sous l'angle financier des questions de répartition des compétences, lesquelles sont déterminantes pour les citoyens concernés,

On ne peut pas, d'un côté, reporter de deux ans toute évolution du schéma financier pour préserver le et, de l'autre, laisser s'affaiblir un acteur central de l'équilibre métropolitain. Je le dis d'autant plus sérieusement et sereinement que la mise en oeuvre de la loi NOTRe aurait bien apporté des recettes supplémentaires à la MGP, grâce notamment à la restitution de la dotation d'intercommunalité, qui est aujourd'hui versée aux EPT.

de province qui ne sont pas forcément rompus aux affaires de la métropole et des établissements publics territoriaux qui ont été créés. Nous sommes confrontés, nous le savons tous, à une réforme bancale, qui ne fonctionne pas très bien, et qui prive régulièrement chacun des échelons de la métropole des crédits nécessaires

de certains établissements publics de coopération intercommunale consécutifs à la contribution au redressement des finances publiques. Dans cette décision, le juge constitutionnel a censuré, dans leur rédaction initiale, les dispositions prévoyant la reconduction annuelle à compter de 2018 et leur caractère figé, qui ne permettait pas une révision du montant prélevé en cas d'évolution « de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés ». Le présent amendement tend simplement à préciser le mécanisme de révision du montant prélevé en cas d'évolution de la situation de la collectivité depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques introduit à l'Assemblée nationale. Il vise notamment à fixer à 5 % le pourcentage de baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant au-delà duquel il sera considéré que la situation du groupement aura évolué de manière suffisamment sensible pour justifier une minoration de son prélèvement sur fiscalité. Ce seuil a été retenu par analogie avec celui qui est pris en compte dans le dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale subies par les collectivités territoriales. Il est enfin prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l'année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021.

qui, en raison des rigueurs de la procédure, ont été déclarés irrecevables. Pourtant, par ces amendements, nous soulevions un réel problème, sur lequel je vais donc me permettre de vous interroger, monsieur le secrétaire Vous savez qu'à la suite de reports, il a été décidé que les plans d'occupation des sols des communes ne seraient plus valables à compter du 31 décembre 2020.

eau, énergie, hydroélectricité, biodiversité, richesse paysagère, etc. La préservation d'espaces naturels de qualité, souvent imposée par le législateur,

à M. Bernard Delcros. En 2019 a été créée la dotation « Natura 2000 ». Cette belle avancée fut une première reconnaissance des aménités apportées par la ruralité, notamment par la montagne. Nous la réclamions depuis longtemps.

mon collègue Claude Raynal a expliqué que les territoires de montagne bénéficiaient déjà d'un certain nombre d'avantages. Ils n'ont donc pas vocation à bénéficier de ce type d'enveloppe.

Les contraintes subies par les communes en raison des zones de protection environnementale ne sont pas forcément liées au nombre d'habitants ; elles sont également liées aux superficies.

Afin de respecter la volonté de la loi, c'est-à-dire de rendre éligibles 60 % des ensembles intercommunaux, il est nécessaire de sortir de ce classement les établissements qui ne sont pas éligibles. C'est pourquoi le présent amendement propose, à compter de 2021, de sortir les ensembles intercommunaux et les communes isolées du classement des entités éligibles au reversement- en fonction de leur indice synthétique de reversement

Cette disposition permettait de faire en sorte que la péréquation soit renforcée pour les communes « pauvres » qui en ont le plus besoin, même si elles font partie d'un EPCI riche. La contribution des communes les plus pauvres au FPIC a été supprimée il y a deux ans. Cependant, la question de l'attribution de financements à ces communes les plus pauvres au titre de la péréquation reste entière.

et compte tenu des moyens financiers, qui sont par essence même toujours limités, il nous faut davantage d'informations pour faire nos choix. Cet amendement vise à demander la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir. Pour autant, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en oeuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. Cette situation s'est aggravée à la suite de la crise sanitaire, ce qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités. La volonté du Gouvernement étant de faire de l'action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d'augmenter le soutien financier de l'État aux collectivités. Or, me semble-t-il, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir si les moyens de fonctionnement et d'investissement sont suffisants et efficients pour mettre en oeuvre les politiques publiques. La vertu d'un rapport demandé au Gouvernement, mes chers collègues, ne doit pas être ignorée ni boudée. Elle permet de lui imposer en quelque sorte un bilan d'étape, de nous le communiquer- normalement -et en somme de nous montrer ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Cela nous permettra de juger comment il répond à l'urgence qui est la nôtre de concrétiser la transition écologique. En la matière, lister ce qui s'est fait, où, pour quels effets, avec quel budget, me paraît capital. Comment progresser dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre sans réaliser des points d'étape, sans regarder avec une grande acuité les efforts consentis et les résultats obtenus ? L'amendement

Or les préfets de département et de région ont l'obligation de publier sur leur site internet les listes de projets financés par la DETR et la DSIL. Les objets sont connus, ce qui permet de savoir exactement à quoi ont servi ces dotations et vers quoi elles ont été fléchées. À mon avis, au-delà de la mission parlementaire, ces amendements sont satisfaits. J'en demanderai donc le retrait.

La séance est suspendue.